monsieur le président.

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement n° 8 rectifié, au sein de l'article 2.

une partie du temps de décharge ne bénéficie pas aux directeurs. Cette situation contribue à rendre plus compliqué l'exercice de leurs missions, puisqu'ils ne sont pas suffisamment déchargés de leur temps d'enseignement. pour rendre attractive la fonction de directeur. Cet amendement vise à organiser une fois par an une présentation de la politique du directeur académique en matière de décharges de temps scolaire et des moyens qu'il mobilise pour que celles-ci soient réellement mises en oeuvre

d'élèves, en pratique, des raisons conjoncturelles peuvent justifier l'utilisation exceptionnelle d'heures de décharge supplémentaires.

Le but de l'article 2 est de faciliter la décharge des directeurs et directrices d'école, qui dénoncent par ailleurs un alourdissement de leur charge administrative. Or, ici, on leur ajoute des missions supplémentaires, ce qui va encore accroître leur charge de travail. De plus, la mission de formation est extérieure au fonctionnement de l'école.

Le texte qui nous est soumis prévoit que, lorsque le directeur exerce sa fonction à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. La mission de formation ne relève aucunement d'un directeur d'école. Nous venons tous de répéter que le directeur était noyé sous des tâches sans cesse plus nombreuses. Ne lui ajoutons pas la formation : le directeur n'est pas un inspecteur. Il doit d'abord se consacrer aux missions de gestion de son école, lesquelles sont multiples et surviennent souvent de façon inopinée : assurer le lien entre les membres de la communauté éducative, gérer les urgences, les mécontentements, les blessures des élèves, les locaux hors d'état, la sécurité, la paperasse ... Et la liste n'est pas exhaustive. Ne trouve-t-on pas que les directeurs ont assez à faire, dans des conditions de décharge et d'exercice de leurs missions souvent très contestables ? Ne chargeons donc pas la barque en leur confiant une nouvelle mission, qui ne relève pas de leurs attributions et qui risque de les placer en porte-à-faux vis-à-vis des enseignants, au corps desquels ils appartiennent. Les directeurs doivent s'occuper de leur école. Cela leur suffit

Monier. Notre amendement tend à préciser que c'est le conseil d'école qui définit le projet pédagogique, et non le directeur, à qui incombe la mission d'assurer ensuite son pilotage. Les attributions du conseil d'école sont prévues dans des articles à valeur infralégislative du code de l'éducation. L'article D. 411-2 définit ainsi ses compétences, dont l'établissement du projet d'organisation pédagogique de la semaine et l'association à l'élaboration du projet d'école, sur proposition du directeur d'école. Nous souhaitons clarifier le texte, qui est quelque peu confus, puisqu'il évoque le pilotage du projet pédagogique par le directeur.

tout au long de la carrière -pour exercer les fonctions de directeur est importante. Cet amendement tend à prévoir que, pour les directeurs d'école en poste, cette formation ait lieu au moins

création d'un corps- tout le monde est d'accord sur ce point -et qu'il s'agit bien d'une fonction que peuvent exercer tous les professeurs des écoles au cours de leur carrière, il semble utile qu'un module sur la fonction de directeur soit proposé lors de la formation initiale des professeurs. Quel est l'avis de la commission

Au vu de leurs très nombreuses tâches et responsabilités, les directeurs d'école doivent pouvoir être assistés par un ou plusieurs agents administratifs. Ces tâches relevant de la compétence de l'éducation nationale, c'est bien à l'État, et non aux communes ou à leurs groupements, de les prendre en charge. Quel

L'article 4, qui prévoit la possibilité pour le directeur d'école de gérer ce temps périscolaire, sous réserve de son accord, avec la collectivité, entraîne une confusion dans la répartition des compétences et des responsabilités qui en découlent entre les collectivités territoriales et l'éducation nationale. Sur ces temps éducatifs périscolaires, la responsabilité reste celle de la collectivité territoriale compétente, y compris si un agent de l'État participait à cette organisation. La collectivité territoriale compétente peut d'ailleurs être différente pour la gestion de l'école et du périscolaire, ce que ne prévoit pas l'article. L'état actuel du droit n'interdit pas aux enseignants, et aux directeurs d'école, de contribuer, de façon contractuelle, à l'organisation et à la mise en oeuvre des temps périscolaires. Cette nouvelle inscription dans la loi irait à l'encontre de la bonne organisation de ces activités à l'échelon local. La

de gérer le temps périscolaire en accord avec la collectivité, est en l'état susceptible de brouiller encore plus les frontières entre l'éducation nationale et la collectivité et d'aller à l'encontre de la bonne organisation de ces activités à l'échelon local. La parole est

: plusieurs régimes d'organisation des activités périscolaires coexisteront selon qu'une convention aura été passée, ou non, entre la commune et le directeur d'école.

de directeurs d'école. Nous avions, dans certaines écoles, un problème d'organisation du temps de restauration. Nous étions alors bien contents de pouvoir nous appuyer sur les directeurs dans un système

perdre toute crédibilité. Enseigner, ce n'est pas seulement rester six heures dans une école. Cela suppose tout un travail de préparation et de prise en charge de la différenciation scolaire pour accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions et leur offrir une éducation à la hauteur de leurs attentes.

n° 13 rectifié . Monsieur le ministre, vous connaissez mon engagement en faveur du développement des instances de participation des jeunes et de la prise en compte de la parole et de l'engagement des jeunes. Je défends, avec trente-sept collègues cosignataires, un amendement de suppression de l'article 4 qui instaure la possibilité de créer un conseil de la vie écolière sur un modèle apparemment proche des conseils de la vie lycéenne ou collégienne, mais dans une école, qui n'est pas un établissement. La volonté de faire toujours plus va parfois à l'encontre de la nécessité de faire bien. Notons-le, la création de ce type d'instance n'était pas interdite avant ce texte et ne sera pas obligatoire après. Cet article ne constitue en fait qu'une recommandation ne créant aucun droit nouveau. Simplement, il tend à rigidifier une composition.

qui est responsable des bâtiments, des aménagements, du périscolaire et du temps méridien. Si ce conseil n'aborde pas ces questions, à quoi s'intéressera-t-il ? De cela, pas un mot dans le texte ! Ce conseil de la vie écolière est en fait une mauvaise idée, dissimulée derrière une bonne intention. Évoquons quelques conséquences de cette éventuelle création. C'est une structure lourde à installer et à animer, une triple élection devant être organisée, sans administration pour le faire. Ce travail reposera donc de fait sur les seules épaules du directeur d'école. créera une confusion avec les missions et les rôles des autres instances existantes, notamment le conseil d'école. La multiplication des instances et des réunions, qui va à l'encontre de la volonté de renforcer la participation des parents dans les conseils d'école,

un tel conseil ne paraît pas approprié par rapport aux attentes éducatives liées à l'âge des enfants en école maternelle ou élémentaire. L'école primaire et maternelle est un lieu d'apprentissage des savoirs fondamentaux de base. Ces savoirs sont un prérequis indispensable à la participation active à une structure telle

amendement tend à préciser que, si le directeur consulte le conseil d'école, il reste le décisionnaire de la mise en place du vote électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves.

risques sont susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. Les directeurs d'école complètent déjà ce PPMS, en lien avec les collectivités compétentes, en fonction des spécificités de l'établissement scolaire, que les inspecteurs et le personnel académique vérifient puis valident. Afin de ne pas introduire une défiance à l'encontre de l'organisation existante, il est nécessaire de maintenir ce travail de préparation commun, qui permet de faire face à tous ces types de situations d'urgence, prévisibles ou non. Cet amendement vise ainsi à garantir un travail plus collaboratif entre le directeur d'école agissant au nom de l'autorité académique et les et les collectivités concernées. De même, l'information du conseil d'école semble être conforme au rôle et aux missions de cette instance, qui réunit la communauté éducative. L'adoption de

et expertes. Tout cela est bien compliqué ! En effet, pourquoi prévoit-on la consultation par les directeurs d'école de personnels compétents en matière de sécurité pour les aider à compléter le plan ? Des personnels compétents en matière de sécurité seront déjà associés à l'établissement du plan par les autorités, en vertu de la deuxième phrase de l'alinéa que nous examinons. Il s'agit donc d'une consultation redondante. Surtout, la consultation de personnels compétents en matière de sécurité par le directeur aura vraisemblablement un coût. le financement de cette charge supplémentaire n'est pas prévu aux termes de la loi. Qui s'en acquittera ? La commune ? L'école ? Sur quel budget ? Nous préférons, compte tenu de ces incertitudes, proposer la suppression de la mention permettant au directeur de consulter des personnels compétents en matière de sécurité, puisque ce sera déjà fait au début de l'élaboration du PPMS.

explication de vote. Je tiens à saluer le travail de M. le rapporteur, notre collègue Julien Bargeton, et de la commission présidée par Laurent Lafon. Le Sénat a été au rendez-vous pour améliorer cette proposition de loi. Les avancées retenues sont attendues par les directeurs et les directrices d'école. Nous avons progressé s'agissant de la reconnaissance, renforcé le cadre juridique, facilité la gestion du temps et la formation.

fonctionnelle et non pas hiérarchique. Il pourra rester un pair parmi ses pairs pour piloter le projet pédagogique et aura les moyens d'assumer les fonctions d'organisation de l'école, en particulier avec ses partenaires.

l'agenda social ouvert, fait que, sur ces questions, il faut bien le reconnaître, des progrès ont été enregistrés. Le groupe Les Républicains votera donc cette proposition de loi.

Résultat des courses, ils auront des missions supplémentaires de formation et de coordination : c'est écrit noir sur blanc ! Des interrogations subsistent pour les directeurs des écoles de moins de quatre classes,

de la proposition de loi. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence,